Nous poursuivons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Enseignement scolaire ».

accélérée des crédits de la loi triennale de programmation. Une observation un peu plus détaillée révèle que vous payez cher un certain nombre de décisions antérieures,

de la qualité des candidats aux concours, notamment dans des disciplines importantes comme le français ou les mathématiques. Vous avez mis fin à cette politique inflationniste, et nous ne pouvons que

de conforter des enseignements traditionnels dont nous pensons, les uns et les autres, qu'ils sont utiles à la formation de nos cadres : je pense en particulier aux langues dites « mortes », qui sont bien vivantes au regard de la déclinaison et de l'explication des concepts d'aujourd'hui

le deuxième cycle du secondaire, c'est-à-dire le lycée. On sent bien, monsieur le ministre, que vous êtes en train d'engager une évolution qui pourrait permettre de s'attaquer aux faiblesses fondamentales

projet de budget, monsieur le ministre, donne clairement la priorité à l'école primaire et à la maîtrise des fondamentaux par tous les élèves. Les savoirs fondamentaux- lire, écrire, compter, respecter autrui -sont la condition de l'acquisition C'est dans les toutes premières années de la scolarité que se joue la réduction de la difficulté scolaire, ainsi que du déterminisme social qui caractérise notre système éducatif. Parce qu'il amorce un rééquilibrage de la dépense d'éducation en direction du primaire, ce budget est un bon budget. Les moyens sont mis au service de la politique éducative, et non l'inverse. C'est pourquoi notre commission a donné un avis favorable à son adoption, sous réserve de l'adoption de l'amendement que je présenterai. J'ai souhaité, monsieur le ministre, concentrer mon propos sur la question du remplacement des enseignants absents. Il s'agit d'un enjeu de confiance à l'égard des élèves et de leurs familles : il n'y aura pas d'école de la confiance sans continuité du service public. Le remplacement des enseignants absents constitue également un véritable défi pour le système éducatif

Dans le premier degré, une absence sur cinq environ n'est pas compensée. Le remplacement y est peu efficient, en raison de la segmentation des remplaçants en brigades spécialisées selon le lieu ou la nature de l'absence à pallier. La circulaire du 15 mars 2017 visait à y remédier, mais son application demeure partielle. Dans le second degré, le remplacement est scandaleusement insuffisant pour les absences de courte durée, au point que la Cour des comptes le qualifie de « défaillance systémique Les protocoles prévus par le décret de 2005 ne sont pas mis en oeuvre ; ils ont été réactivés dernièrement par une circulaire, mais celle-ci ne crée pas pour autant les conditions de leur application effective. Cette situation pourrait encore s'aggraver du fait de la pénurie d'enseignants dans de nombreuses académies, qui impose un recours accru aux contractuels. L'enseignement privé connaît une situation critique du fait de l'écart de rémunération entre ses remplaçants et ceux du service public. Un alignement des rémunérations me semble nécessaire. Mes chers collègues, le remplacement est un problème non pas de moyens, mais d'organisation du service, qui révèle l'urgence d'une réflexion d'ensemble sur la gestion des ressources humaines du ministère.

Le remplacement des collègues absents et la formation continue doivent être intégrés aux missions des enseignants. Je recommande également l'annualisation des obligations de service et le développement de la bivalence dans le second degré. Enfin, j'observe que l'éducation, premier investissement de la Nation, est paradoxalement peu présente dans cet hémicycle. La politique éducative mérite mieux qu'une soirée consacrée à l'examen de ses crédits. C'est pourquoi je souhaiterais que se tienne chaque année au Sénat, avant les arbitrages budgétaires, un débat d'orientation sur les politiques d'éducation. Très bien ! Le Parlement doit se saisir de ce sujet décisif pour l'avenir de notre pays et dont le Président de la République a fait une priorité. J'espère, monsieur le ministre,

égalité de traitement avec l'éducation nationale témoigne de la priorité accordée par le Gouvernement à l'éducation et à la formation professionnelle. Notons toutefois que ce budget ne prend pas en compte l'évolution probable des subventions aux établissements privés, qui accueillent plus de 60 % des élèves de l'enseignement agricole. Les protocoles actuels qui, par dérogation avec la loi Rocard, plafonnent le montant des subventions versées expireront le 31 décembre prochain. Pour l'enseignement privé du temps plein au moins, les négociations sont en cours, les fédérations exigeant à ce stade une revalorisation substantielle, demande à laquelle le ministère doit apporter une réponse. Je forme le voeu que ces négociations aboutissent. Composante essentielle de l'enseignement agricole, le secteur privé mérite un traitement équitable. J'ai l'intime conviction que cette filière de réussite et d'excellence a de l'avenir. Alors qu'il existe une demande et un véritable besoin dans certains territoires, en particulier à Mayotte et en Guyane, mais aussi dans certains départements de la France hexagonale, l'enseignement agricole doit sortir d'une logique de conservation pour entrer dans une dynamique d'expansion. Il s'agit d'atteindre un objectif ambitieux : offrir une formation de qualité à la jeunesse et soutenir, par la formation, le développement de l'agriculture, secteur clé pour de nombreux territoires, notamment en outre-mer.

malgré ses résultats enviables en matière d'insertion professionnelle, bien supérieurs à ceux de l'éducation nationale. Les effectifs de l'enseignement agricole baissent de manière continue depuis 2008, à rebours des évolutions démographiques. Cela s'explique en grande partie par la dévalorisation de l'enseignement agricole dans les représentations, ainsi que par la réticence de l'éducation nationale à orienter les élèves j'appelle de mes voeux le lancement d'une grande campagne de promotion associant l'éducation nationale et visant à mettre en avant les réussites de cet enseignement et la diversité des formations et des métiers auxquels il prépare.

Celle-ci pourrait être utilement renforcée en matière d'orientation, d'élaboration de la carte des formations, de formation initiale et continue des enseignants, de remplacement et d'accompagnement des élèves en situation de handicap. En matière tant de formation professionnelle que d'intégration de l'alternance ou de résorption de la difficulté scolaire, l'enseignement agricole est une filière exemplaire et riche, et son développement

... Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

Si nous avons bien compris, ce projet de budget est bâti selon le schéma dominant suivant : une école efficace pour que chaque élève, à la fin du primaire, sache lire, écrire et compter, ainsi que respecter autrui.

L'orientation actuelle, qui consiste à relancer les classes de latinistes ou d'hellénistes, ou encore les classes bilangues, pour quelques-uns seulement, plutôt que d'enseigner une seconde langue dès le plus jeune âge, nous interpelle. L'efficacité scolaire est-elle toujours une garantie de l'équité ? Une école efficace est-elle aussi celle du bien-être et du développement de l'autonomie des élèves ?

avec des maîtres spécialisés pour des enfants en difficulté, ont montré qu'une diminution des effectifs n'était pas toujours une réponse suffisante pour remédier efficacement aux problèmes des élèves, et que les méthodes et le choix des enseignants comptaient aussi. Pour ces raisons, nous devons donc maintenir la formation que certains de vos prédécesseurs avaient supprimée. Nous craignons que, pour dédoubler les classes, on assèche le dispositif « Plus de maîtres que de classes » mis en place auparavant et plébiscité par les enseignants.

Nos craintes paraissent d'autant plus fondées que le projet de budget que vous nous soumettez, monsieur le ministre, porte un coup d'arrêt au recrutement dans le premier degré. Le nombre de postes ouverts aux concours d'entrée dans le métier d'enseignant se resserre dès l'année prochaine.

Par ailleurs, laisser aux acteurs le choix de conserver la semaine de quatre jours et demi ou de revenir à quatre jours ne nous semble pas aller dans le sens de l'intérêt des enfants. Toutes les études que nous avons consultées à ce sujet soulignent combien la concentration des apprentissages sur quatre jours est néfaste pour les enfants, surtout pour les plus défavorisés d'entre eux, qui sont aussi ceux dont les activités périscolaires sont le plus erratiques. L'OCDE avait pourtant noté que la réforme des rythmes éducatifs allait dans le bon sens. Certes, vous n'interdisez pas la semaine scolaire sur neuf demi-journées et vous maintenez les dotations qui s'y rapportent,

Le montant des autorisations d'engagement prévues pour les actions éducatives complémentaires aux enseignements et pour la vie scolaire est plutôt de nature à nous inquiéter. En marge du débat budgétaire, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de fixer enfin, après une large consultation, une semaine scolaire qui convienne réellement au rythme des enfants des écoles de notre pays ? Il n'est pas sain de laisser les intérêts économiques et les influences les plus diverses modeler le fonctionnement de nos écoles. Si, dans le secondaire, une mesure comme la mise en place du dispositif « Devoirs faits » nous semble juste et conforme aux réformes engagées auparavant, nous nous demandons en revanche si les budgets nécessaires à un accompagnement efficace sont toujours au rendez-vous. au numérique est également indispensable pour que notre système éducatif se mette à l'heure du XXI siècle. En 2017, un important effort a été réalisé dans ce domaine, notamment dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, mais l'on ne voit pas ce qui est prévu pour continuer dans ce sens en 2018. La grande oubliée de ce projet de loi de finances est la médecine scolaire. Voilà des années que nous avons du mal à faire face à une crise sanitaire qui s'aggrave. Aujourd'hui, nous savons que les postes n'ont pas été pourvus parce que la situation des médecins scolaires n'est pas suffisamment attrayante en termes de revenus, d'indemnités, de prise en charge des frais.

Avant de conclure, je dirai quelques mots sur les crédits du programme 143 « Enseignement technique agricole », qui sont en augmentation de 2,5 %.

l'on sait que 80 % des jeunes qui s'installent en agriculture ne sont pas originaires du monde agricole, on mesure mieux la réussite de l'enseignement agricole en termes d'insertion professionnelle. Monsieur le ministre, les sénateurs du groupe socialiste et républicain demeureront très vigilants sur les améliorations qu'il convient d'apporter à ce projet de budget qui, pour le moment, s'agissant de ses orientations,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'enseignement scolaire est un sujet fondamental pour l'examen du projet de loi de finances pour 2018. Notre pays compte plus de 12 millions d'élèves scolarisés : près de 7 millions dans le premier degré et près de 6 millions dans le second. Pour prendre en charge ces élèves, pas moins de 875 000 enseignants sont mobilisés chaque année, tous secteurs confondus, dans le système scolaire. En matière d'éducation, nombre d'hommes politiques parlent, mais peu agissent vraiment. Notre nouveau ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déjà su démontrer qu'il était un homme d'action. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, vous trouverez sur nos travées des soutiens de votre politique. L'éducation n'est pas un sujet politique comme les autres ; c'est un enjeu de formation des générations futures, puisqu'il s'agit d'instruire les jeunes élèves pour en faire des citoyens. 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République avait pour ambition de remettre à plat le système scolaire français. Ses dispositions tendaient à réformer l'enseignement du socle commun de connaissances, à accroître les connaissances et les compétences culturelles de nos têtes blondes, à assurer la lutte contre les inégalités sociales et territoriales et à améliorer la réussite de nos élèves. Le précédent gouvernement, à l'origine de ce texte, nous avait promis un système éducatif juste et efficace dans l'accès au savoir. En étant extrêmement charitable, le moins que l'on puisse dire est que ces ambitions n'ont pas été atteintes, bien au contraire Le système scolaire français est vieillissant, parfois même inopérant. Il traverse une crise profonde. Ainsi, les niveaux de performance des élèves français en mathématiques se sont dégradés de manière importante entre 2003 et 2012 et stagnent depuis le niveau global des élèves français en sciences se situe en deçà des moyennes européenne et internationale. La proportion des élèves en difficulté scolaire est passée de 21 % en 2006 à 22 % en 2015, celle des élèves en échec scolaire de 15 % en 2004 à 20 % en 2013. Enfin, les élèves issus de milieux défavorisés ont quatre fois plus de risques de souffrir de difficultés scolaires, contre trois fois en moyenne dans les pays de l'OCDE, atteste la fin de l'égalité des chances à l'école. C'est un constat pénible à dresser, mes chers collègues, d'autant que l'enseignement scolaire touche à l'avenir de notre pays et au bien-être des familles françaises. C'est dans les premières années de scolarité que notre école forme l'enfant à devenir un citoyen honnête et un travailleur sérieux. Il faut donc réaffirmer la priorité donnée à l'enseignement de premier degré, notamment à la scolarisation des enfants de moins de trois ans ; c'est ce que vous avez décidé de faire, Il faut aussi soutenir nos enseignants, par exemple en renforçant le remplacement pour formation continue des maîtres. Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » va dans le bon sens, et nous le soutenons. Il s'agit de réduire les inégalités en apportant une aide renforcée aux populations scolaires les plus fragiles. Cette mesure prévoit l'affectation d'un enseignant supplémentaire au sein d'une école ou d'un groupe scolaire pour mieux répondre aux besoins des élèves

D'autres mesures, lancées sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, nous invitent à garder espoir en un avenir plus radieux. Les choses peuvent encore changer dans notre système scolaire le dédoublement des classes de CP et CE1 à douze élèves dans les quartiers défavorisés, promesse faite par le futur Président de la République pendant la campagne présidentielle, s'est appliqué à la rentrée 2017 pour 2 200 classes de cours préparatoires, 2 500 postes ont été attribués pour accompagner les écoles des réseaux d'éducation prioritaire et des réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Cette initiative s'inscrit dans la feuille de route du ministère en vue de réduire les inégalités entre les familles.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement assure que les années 2017 et 2018 seront déterminantes dans la refondation de notre système d'enseignement scolaire. Les sénateurs du groupe Les du groupe Les Indépendants l'espèrent ! Ils voteront les crédits de la mission, tout en formulant plusieurs propositions pour que les dispositifs déployés par le nouveau Gouvernement soient analysés rapidement et fassent l'objet d'une évaluation dès que possible.

monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de budget donne la priorité à l'enseignement primaire. Les membres du groupe du RDSE saluent ce recentrage. La maîtrise des fondamentaux demeure en effet la clef de la réussite scolaire, ainsi que le principal moteur de l'émancipation individuelle de nos élèves. La création de 2 800 postes supplémentaires est prévue pour mettre en oeuvre le dédoublement des classes de CP et de CE1 au sein des écoles REP et REP+. Il conviendra toutefois de veiller à ce que cette importante mobilisation ne conduise pas aussi à un nouvel assèchement du vivier de remplaçants au sein de l'enseignement primaire. si la question de la maîtrise des fondamentaux est essentielle, celle du non-remplacement d'un grand nombre d'enseignants dans un délai raisonnable, notamment pour les courtes absences, est toujours particulièrement préoccupante. Le déploiement de ce nouveau dispositif impliquera également d'importants aménagements en termes de bâti scolaire. Une part des 615 millions d'euros de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, de finances, doit y être affectée, afin d'accompagner les collectivités territoriales dans cette nécessaire adaptation. Dans un schéma d'emplois que vous avez voulu neutre, ces nouvelles créations de postes dans l'enseignement primaire se feront aux dépens de 2 600 postes d'enseignants stagiaires dans le secondaire, qui seront supprimés. Là encore, la vigilance s'impose sur les signaux que nous envoyons, alors que se poursuit la crise du recrutement des enseignants, une profession réputée difficile et mal rémunérée au regard des études demandées. Le corps enseignant est d'ailleurs en attente d'une revalorisation de son traitement annoncée- réforme Parcours professionnels, carrières et rémunérations et prime aux enseignants en REP+ -, mais dont la mise en oeuvre se fait toujours attendre. Le manque d'attractivité de la profession conduit, année après année, à multiplier le recours à des contractuels de plus en plus précaires. Par ailleurs, des milliers de candidats sont recrutés chaque année sans avoir la formation d'enseignant, ni même, souvent, la connaissance la plus élémentaire de la discipline enseignée. concerne l'enseignement agricole, les efforts consentis en faveur de l'enseignement primaire n'ont pas de conséquences en termes de suppressions de postes. Les effectifs demeureront stables, après plusieurs années de hausse. Il convient de saluer l'excellence de l'enseignement agricole français, dont les taux d'insertion professionnelle sont tout à fait remarquables, et ce avec une part d'élèves boursiers supérieure à celle observée au sein de l'éducation nationale. Pourtant, en dépit de ces excellents résultats, l'attractivité de l'enseignement agricole va s'estompant. Les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture doivent s'employer à revaloriser l'image des filières agricoles et à accroître la visibilité de cette orientation. Le groupe du RDSE se félicite aussi de la forte augmentation que connaissent les crédits consacrés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Cette hausse, de 46 %, doit permettre le recrutement d'accompagnants et la poursuite de la professionnalisation Je conclurai mon propos en évoquant la situation de la médecine scolaire, à la suite d'autres orateurs. On recense actuellement, en moyenne, un médecin scolaire pour 12 000 élèves. Les rémunérations et les diverses prises en charge allouées par l'État sont insuffisantes pour assurer une réelle attractivité de ces postes. Les politiques de santé publique conduites en milieu scolaire s'en ressentent nécessairement. Comme nous le savons, s'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, des troubles auditifs ou visuels peuvent représenter un obstacle majeur à l'épanouissement et à la réussite scolaire. Les politiques de prévention en matière sanitaire jouent également un rôle très important. Les difficultés rencontrées pour rétablir une médecine scolaire adaptée sont croissantes depuis plusieurs années, et force est de constater que ce projet de loi de finances n'apporte pas de réponse à cette préoccupante dégradation. Le suivi médical des enseignants au cours de leur carrière peut d'ailleurs faire l'objet du même constat : s'il y a bien une visite médicale lors de l'embauche, aucune

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il nous est proposé de porter les crédits de la mission interministérielle « Enseignement scolaire » à 71,5 milliards d'euros de crédits de paiement qui représente 25,68 % du budget de l'État. Près de 93 % de ces crédits sont destinés à des dépenses de personnel. termes, la mission de l'État dans ce domaine ne consiste plus qu'à payer les enseignants placés devant les élèves. Ce rôle exclusif sera accentué par ce projet de budget, qui poursuit le désengagement dans la médecine scolaire, supprime 200 postes dans la filière administrative et menace le financement des manuels scolaires. Il faut donc garder à l'esprit que tout le reste est à la charge des collectivités Il eût été intéressant d'évaluer, pour mémoire, toutes les dépenses qu'elles assument pour assurer le service public de l'éducation nationale, tant en fonctionnement qu'en investissement. comprennent notamment l'entretien et la gestion des bâtiments, mais aussi, par exemple, la restauration et le transport scolaires. Pour tout cela, il n'y a plus d'égalité de traitement entre les familles, et les disparités entre collectivités territoriales sont très importantes. Je prendrai un seul exemple il n'y a pas de ramassage scolaire dans les départements très urbains de la métropole parisienne, alors que cette dépense peut être considérable dans les départements ruraux. Elle représente aujourd'hui plus 3 milliards d'euros, et de nombreuses collectivités territoriales ont décidé d'en faire supporter une partie du coût aux familles. donc conscience ensemble que l'accès au service public de l'éducation nationale est de moins en moins gratuit et de plus en plus territorialement inégalitaire.

de l'évolution positive de la démographie. Cette hausse concerne essentiellement les dépenses du titre 2, c'est-à-dire la masse salariale. La loi de programmation des finances publiques prévoit un net ralentissement de cette augmentation pour les années à venir. Disons-le avec force : après les tentatives de rattrapage du gouvernement précédent, l'actuel gouvernement organise une nouvelle diminution des emplois d'enseignants à partir de 2019, ce dont se félicite d'ailleurs le rapporteur spécial, M. Longuet. Absolument ! Le projet de budget pour l'année 2018 n'est donc qu'une parenthèse de stabilité dans un processus de décroissance à venir. J'utilise à dessein le mot « stabilité », car l'examen attentif du projet de budget fait clairement apparaître que l'essentiel de la hausse acceptée pour 2018 concerne des mesures liées à l'augmentation de la masse salariale entre 2012 et 2016. Elle résulte de la création d'environ 35 500 nouveaux postes sur les 55 000 postes prévus par la loi dite « d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ». termes, il n'y a plus de création nette d'emplois à espérer pour 2018 et les années suivantes. Les dispositifs nouveaux devront être organisés par le biais de redéploiements de postes. Ainsi, l'effort indéniable en faveur de l'enseignement primaire est réalisé uniquement grâce à la suppression d'environ 2 600 postes d'enseignants dans le secondaire et 2 100 postes d'enseignants stagiaires. utilisant un mot employé pour d'autres ministères, il faut donc constater que le Gouvernement a décidé de contenir absolument le « format » de l'éducation nationale. est d'ailleurs le constat du rapporteur spécial, qui fait observer : « La logique quantitative poursuivie sous le précédent quinquennat semble avoir été abandonnée par l'actuel gouvernement au profit d'une gestion plus raisonnée des effectifs ». Il faut entendre par cette délicieuse formule qu'il n'y aura plus de créations de postes et qu'il faudra faire autant, ou plus, avec moins. Nous entrons donc de nouveau dans une période de gestion de la pénurie,

qu'il existe un lien fort entre le nombre d'élèves par classe et les résultats scolaires et dédoublez en conséquence les classes de CP des réseaux d'éducation prioritaire renforcés ; mais, dans le même temps, vous faites porter l'essentiel de la charge de ces mesures nouvelles sur l'augmentation du nombre d'élèves par classe dans les collèges et les lycées. Cette politique de transfert est d'autant plus préoccupante que l'arrivée de 30 000 élèves supplémentaires est prévue dans les collèges et que de nombreuses classes de lycée présentent aujourd'hui, dans certaines académies, des effectifs supérieurs à Par ailleurs, on peut légitiment s'interroger sur votre capacité à mettre en oeuvre vos nouveaux dispositifs d'accompagnement des élèves dans un cadre d'emplois aussi contraint et avec la disparition des emplois aidés. Le risque est sans conteste d'assister de nouveau à une dégradation majeure des conditions d'enseignement. Ce n'est pas une bonne chose pour l'éducation nationale, qui doit affronter une grave crise des vocations. cette année, à l'issue du concours du CAPES, quelque 374 postes n'ont pas été pourvus pour l'enseignement des mathématiques, ni 343 pour celui de l'anglais, ni 220 pour celui de l'allemand ? Je finirai cette triste énumération par les lettres classiques, pour lesquelles 63 % des postes ouverts au concours n'ont pas été pourvus ... Dans un contexte de chômage élevé et de réduction des débouchés pour les diplômés de l'enseignement supérieur, cette désaffection est la conséquence de l'appréciation négative portée par la jeunesse sur le métier d'enseignant et les conditions salariales et matérielles de son exercice. Comme les années précédentes, cette baisse structurelle des emplois statutaires sera compensée par un recours accru aux emplois contractuels, qui atteint dans l'éducation nationale des proportions alarmantes et sur lequel la commission des finances a fort opportunément demandé à la Cour des comptes d'enquêter.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'enseignement scolaire est l'avenir de notre pays. Or chacun sait que nous pourrions mieux le préparer. Depuis plusieurs années, l'école primaire va mal, ce dont témoignent les évaluations de la maîtrise des savoirs fondamentaux par les élèves. Comme le souligne notre rapporteur spécial, à leur entrée en sixième, quelque 82,1 % des élèves maîtrisent les compétences de socle 1, qui portent sur la compréhension d'un texte et les notions élémentaires de vocabulaire, grammaire et orthographe. Ce qui signifie,, que près de 18 % des élèves n'ont pas atteint ce niveau à leur entrée dans le secondaire. Ce chiffre doit être mis en perspective avec un autre, d'ordre budgétaire : le le coût d'un lycéen français est de 38 % plus élevé que le coût moyen d'un lycéen dans les autres pays de l'OCDE. En d'autres termes, nous dépensons trop pour le secondaire, pas assez pour le primaire. Et cette dépense n'est pas efficiente, puisque les efforts consentis pour le collège et le lycée ont bien du mal à rattraper les retards accumulés en primaire. Ce constat est connu et partagé, mais nous avons tardé à en tirer les conséquences. Il semblerait que le présent budget engage une inflexion en ce sens. Il amorce en effet le nécessaire rééquilibrage budgétaire entre primaire et secondaire. Les crédits consacrés au primaire sont en hausse de 2,3 % et 2 800 postes d'enseignants sont créés pour la rentrée 2018, 2018, en contrepartie de la suppression de 2 600 postes d'enseignants stagiaires dans le second degré et de 200 postes de personnels administratifs. Les effets de ce rééquilibrage des moyens seront accentués par l'évolution démographique, la baisse des effectifs d'élèves dans le premier degré renforçant mécaniquement les effets bénéfiques de la mesure.

Nous ne pouvons que soutenir très fortement cette orientation, étant donné surtout que, selon le programme international pour le suivi des acquis des élèves, la France est le pays où les résultats sont le plus fortement corrélés avec le niveau socio-économique et culturel des parents. Le rôle de la puissance publique est de casser le cercle vicieux de la prédestination sociale. Dans la même logique, nous soutenons également la relance des stages de réussite pour les élèves les plus fragiles à leur sortie du primaire, ainsi que le rétablissement des évaluations diagnostiques en CP et à l'entrée en sixième. En ce qui concerne le secondaire, nous comprenons bien que le collège et le lycée devraient faire l'objet de réformes ultérieures. Toutefois, comme nombre de nos collègues, nous déplorons la réduction des crédits en faveur des manuels scolaires au collège. Nous soutiendrons donc vivement l'amendement de notre commission visant à allouer 50 millions d'euros supplémentaires à ce poste, pour éviter que cette charge ne retombe sur les départements, dont les finances sont extrêmement contraintes, alors même que l'État s'était engagé à compenser intégralement le coût induit par la réforme des programmes.

budget maintient les aides du Fonds de soutien aux activités périscolaires en faveur des communes ayant conservé une semaine comptant cinq matinées d'enseignement à l'école primaire. Dernière orientation positive, que nous ne pouvons que saluer : la notable augmentation des crédits consacrés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap, qui permettra de financer le recrutement d'accompagnants et la poursuite de la professionnalisation

scolaire. En réalité, le Gouvernement ayant donné la priorité au primaire, les crédits du secondaire généraliste stagnent. L'enseignement agricole échappe à cette stagnation, ce qui concrétise l'accent mis par le Gouvernement sur la formation professionnelle. Nous ne pouvons que saluer cette consolidation, d'autant que les résultats de l'enseignement agricole en termes d'insertion professionnelle sont très supérieurs à ceux de l'éducation nationale. Le modèle de l'enseignement agricole doit, sans mauvais jeu de mots, faire école. Je pense en particulier aux établissements privés, qui accueillent la majorité des élèves, et, encore plus spécifiquement, aux maisons familiales rurales, les MFR, dont l'enseignement est fondé sur l'alternance.

Leur plafonnement ne doit pas contribuer au déclin des effectifs. Ce serait là un échec regrettable. Tout en restant attentif à l'aboutissement des négociations en cours sur ce sujet, le groupe Union Centriste est favorable aux crédits de la mission « Enseignement scolaire », », contrairement aux années précédentes. Ce soutien, destiné à saluer la rupture que semble initier le présent budget, n'est pas pour autant un blanc-seing donné au Gouvernement. les plus gros chantiers sont à venir, et l'inflexion donnée aujourd'hui ne pourra porter ses fruits que si des réformes de structure, destinées à réaliser des gains d'efficience, sont entreprises dans les années à venir.

dont je salue le travail excellent, à l'annualisation du temps de travail des enseignants, ou encore à l'évaluation de toutes les matières et options, souvent facultatives, très consommatrices en moyens humains et financiers.

Bref, de tout ce qui participe à l'élévation de nos élèves en leur demandant travail et exigence. Ceux-là pensent que baisser le niveau permettra à chacun de réussir et de mieux s'impliquer dans la société actuelle ... Quelle erreur ! Ce qu'ils veulent supprimer, ce sont des marqueurs d'exigence pour nos élèves et leurs parents.

Certains franchissent allègrement la ligne blanche, comme Sud Éducation 93, qui propose des formations non mixtes destinées aux enseignants en stage pour analyser le racisme d'État ... Je sais, monsieur le ministre, que vous avez condamné

Pour la première fois, la dotation de l'enseignement scolaire dépasse le seuil des 50 milliards d'euros. Il convient d'y ajouter le budget consacré à la jeunesse et à la vie associative pour plus de 500 millions d'euros, ce qui représente un budget total de 50,6 milliards d'euros.

La priorité sur l'école primaire, le dédoublement des classes de cours préparatoire dans les zones d'éducation prioritaire, le programme « Devoirs faits », les stages de réussite sont autant d'actions mises en place, dont nous pouvons être fiers. Je tiens à saluer la volonté du Gouvernement d'honorer ses engagements et de tracer un cap vers une école de la confiance, inspirée par trois mots : République, excellence et bienveillance. Nous devons garantir la réussite de 100 % des élèves à l'école primaire. En effet, aujourd'hui, plus de 20 % des élèves sortent de l'école primaire sans savoir correctement lire, écrire ou compter, et ces difficultés concernent plus particulièrement les enfants issus de milieux défavorisés.

Nous devons faire en sorte que chaque élève quitte l'école primaire en maîtrisant la lecture, l'écriture et les chiffres, et qu'à cette période de sa scolarité, il ait acquis la compétence indispensable qu'est le respect. Cette lutte se fera à la racine de la difficulté scolaire, dès les premières années de la scolarité donc. Nous devions agir tout de suite. Aussi, depuis le mois de septembre, le nombre d'élèves en cours préparatoire en réseau d'éducation prioritaire renforcée, REP+, a été limité à Une fois de plus, l'action a succédé à l'engagement du Président de la République. Le projet de loi de finances pour 2018 poursuit cette action et, à terme, plus de 11 000 classes de CP et de CE1 seront concernées. Dans une note de septembre 2017, l'institut des politiques publiques relevait que les effets d'une telle mesure « sont élevés, si on les compare à d'autres politiques scolaires menées à grande échelle et rigoureusement évaluées. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Sans l'acquisition de ces fondamentaux, comment construire sa vie professionnelle, comment vivre pleinement sa citoyenneté ? Par ailleurs, l'école est un incubateur, un révélateur de talents. Elle doit permettre à chaque élève de déceler et cultiver celui qui est le sien. C'est ainsi que l'on atteint sa propre excellence. Pour ce faire, des réponses éducatives adaptées aux réalités du terrain et aux besoins des élèves doivent être apportées. Des moyens sont dégagés dans le projet de loi de finances pour 2018 pour donner davantage de libertés aux communautés éducatives, pour que les acteurs de terrain disposent de leviers plus nombreux pour innover et répondre le mieux possible aux besoins des élèves, notamment sur les rythmes scolaires. Cette liberté donnée et cette confiance témoignée envers les professeurs et les personnels se traduiront également par un soutien constant de l'institution dans l'exercice de leurs missions et dans leurs initiatives. Depuis la rentrée 2017, les établissements et les enseignants bénéficient de marges de manoeuvre accrues, en échange desquelles ils font l'objet d'une évaluation et auront à se responsabiliser dans le cadre de contrats d'objectifs liant les établissements publics locaux d'enseignement et les autorités académiques. C'est dans cet esprit que la réforme du collège a été assouplie à la rentrée 2017. Les parents doivent avoir confiance dans les communautés éducatives, dans les formations qu'elles dispensent et, bien sûr, dans les formations dont elles disposent. Je me permets de mettre l'accent sur la formation qui est, selon moi, la clef de voûte de tout bon système éducatif. La formation des professeurs joue un rôle crucial pour relever le défi auquel la France fait face. Elle doit se caractériser par une entrée plus progressive dans le métier, grâce notamment au développement des formules de prérecrutement. Par ailleurs, la formation initiale et la formation continue ont vocation à se nourrir davantage des apports de la recherche de haut niveau reconnue internationalement et de l'expérience des praticiens. Le projet Enfin, l'école doit être bienveillante et personnaliser le parcours de chaque élève. Le programme « Devoirs faits » en est un exemple. Il permettra aux collégiens de trouver un accompagnement et une aide face aux difficultés rencontrées durant les révisions et des exercices d'approfondissement. Pour conclure, le présent projet de budget traduit l'engagement du Président de la République et de la majorité en faveur de la jeunesse de notre pays. Surtout, et c'est essentiel, il est destiné à lutter concrètement contre l'échec scolaire. Il engage les transformations indispensables pour faire émerger l'école de la confiance qui construira l'avenir de notre pays. C'est le coeur de notre redressement et de notre rayonnement. Bien entendu, le groupe La République En Marche soutient totalement votre action, monsieur le ministre.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation

J'essaie simplement de faire référence aux pays qui vont bien en ce moment, aux pays dont les systèmes scolaires connaissent la réussite et qui ont réussi à bâtir une « école de la confiance », expression que vous avez été plusieurs à reprendre et qui représente en effet la clef de la réussite d'un système. système. Une école fonctionne lorsque la société a confiance en elle et lorsque l'école à son tour produit de la confiance. Pour produire de la confiance, il faut évidemment un budget solide- je crois que ce budget est solide de le montrer -, mais il faut aussi que ce budget corresponde à des objectifs qualitatifs. Le premier de ces objectifs qualitatifs, vous le savez, c'est de donner les savoirs fondamentaux à tous les élèves à la sortie de l'école primaire. Si nous n'atteignons pas cet objectif, nous ne réussirons pas le reste. Cette après-midi, j'assistais en Sorbonne à une conférence appelée « Les Controverses de Descartes », où il était justement question de cet accès aux savoirs fondamentaux et de la qualité des apprentissages.

C'est pourquoi la première caractéristique de ce budget est la priorité donnée à l'école primaire : lire, écrire, compter et respecter autrui sont les quatre piliers du primaire. Derrière cette priorité budgétaire, il existe un volontarisme pédagogique. L'objectif est d'attaquer la difficulté scolaire à la racine. Vous êtes plusieurs à l'avoir rappelé : c'est le sens du dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Après 2 500 classes dédoublées cette année, nous souhaitons en dédoubler 6 000 autres au cours de la rentrée scolaire 2018. Ce sera l'année la plus importante pour l'accomplissement de cet engagement présidentiel.

elle s'accompagne d'une action attentive et qualitative vis-à-vis des écoles rurales. Avec le sénateur Alain Duran, qui s'est impliqué dans l'analyse des contrats départementaux que nous signons en la matière, je me suis engagé

Nous voulons accompagner les élèves vers la réussite dans tous les territoires, qu'il s'agisse des territoires urbains, des territoires dits « périphériques » ou des territoires ruraux.

Je discuterai avec les organisations syndicales au cours des prochains mois pour déterminer les conditions exactes de la mise en oeuvre de cette disposition. Accompagner les élèves vers la réussite passe d'abord par l'école primaire, mais cet objectif se poursuit évidemment avec le collège.

et cela sur une base qui permette d'atténuer, voire de diminuer de façon décisive les inégalités liées au milieu familial. C'est pourquoi une enveloppe budgétaire considérable de l'ordre de 220 millions d'euros

Aujourd'hui, si l'on veut de la mixité sociale, si l'on veut que les collèges ruraux et les collèges de banlieue attirent de nouveau les élèves, il convient de prendre des initiatives de ce type. J'ai fréquemment visité des collèges qui avaient réussi dans nous avons su prendre des mesures spécifiques. C'est par la différenciation, grâce au projet éducatif de chaque établissement, et par notre capacité à donner davantage aux établissements les plus fragiles, que nous réussirons à diminuer les inégalités sociales

De même, l'école inclusive va évidemment faire des progrès à la faveur de ce budget. L'accueil des élèves en situation de handicap est une priorité, partagée par les différentes majorités. Il nous faut mener des actions de long terme sur cette question.

à la cohérence entre ce que nous faisons en matière de savoirs fondamentaux et ce que nous faisons en matière d'ouverture vers d'autres disciplines, notamment par l'éducation artistique et culturelle, par le déploiement à venir des activités périscolaires

afin de donner à cette filière toute l'importance qu'elle mérite. Sur le fond, il faut redonner symboliquement de la valeur à l'intelligence des interactions de la main, de l'outil et de la matière. Pratiquement, nous pensons qu'il est nécessaire de mieux accompagner les élèves des filières techniques et les bacheliers techniques vers des formations supérieures adaptées à leurs besoins, tout en refusant de considérer que, pour eux, l'apprentissage serait la seule voie possible. On ne peut notamment continuer d'accepter que ces bacheliers échouent dans de fortes proportions à entrer dans les instituts universitaires de technologie pour, ensuite, s'égarer dans des formations généralistes qui ne leur sont pas toujours destinées et pour lesquelles ils participent au fort taux d'échec en licence. La résorption de l'encombrement de certaines filières dites « en tension » peut plus justement être trouvée dans le développement de nouvelles formations supérieures pour ces élèves. Cet effort d'adaptation doit nécessairement être entrepris dès le cycle du second degré. S'agissant de l'enseignement agricole, nous regrettons amèrement les fortes difficultés budgétaires auxquelles il est confronté et qui vont encore empirer avec le projet budgétaire pour l'année 2018. Le réchauffement climatique, la protection de l'environnement et les nécessaires mutations des systèmes de culture rendent indispensables de lourds investissements dans la recherche et la formation des agriculteurs. Ces efforts doivent être engagés dans le cadre de l'enseignement agricole. Ils seront effectivement d'autant plus efficaces s'ils s'adressent aux plus jeunes. Par ailleurs, il est grand temps de corriger les distorsions de statut qui isolent les corps de l'éducation agricole. Je pense aux assistants d'éducation de l'enseignement agricole, mais aussi à tous ces postes à responsabilités qui mériteraient d'être accueillis dans des corps plus amples

à affirmer un choix philosophique au profit de l'école laïque et républicaine, que nous revendiquons et que nous assumons. Cette école est la seule qui accueille encore les élèves sans aucune sélection, qu'elle soit sociale, économique monsieur le ministre, toute la justesse de ma remarque sur les valeurs ! Cette mission de service public est d'autant plus difficile à exercer que les quartiers sont en difficultés, car les ghettos sociaux sont aussi des ghettos scolaires. À défaut de pouvoir réduire la ségrégation sociale, notamment par une politique du logement correctrice, l'État doit apporter plus à celles et ceux qui ont moins. notre amendement devrait ainsi permettre de financer, dès 2018, le dédoublement de toutes les classes des réseaux d'éducation prioritaire et l'accueil des élèves pour les devoirs du soir. devoirs du soir. Il nous semblerait juste que les crédits accordés aux institutions privées soient attribués en fonction des charges de service public que celles-ci assument, notamment pour l'accueil des élèves des familles les plus défavorisées. Dans ce domaine comme dans de nombreux autres, il ne serait pas inepte, au moins, de connaître l'utilité sociale d'aides financées par l'impôt citoyen.

un assaut de bonnets rouges bretons ! Je voudrais dire à mon collègue Pierre Ouzoulias que je suis pour la paix scolaire : l'enjeu qui nous préoccupe tous, c'est la réussite de tous les enfants et l'égalité des chances

J'invite donc mon collègue à un stage en Bretagne. J'aurai grand plaisir à lui faire découvrir ce qu'est l'enseignement privé sur notre territoire et ce qu'est la diversité

mais cette attractivité n'a strictement rien à voir avec une espèce de crise mystique. Loin de là ! Ce que souhaite l'immense majorité des parents d'élèves

On peut toujours vouloir plus de moyens, mais il me semble que la crise de l'éducation nationale vient bien plus du dogmatisme idéologique qui l'a hypnotisée, guidée et emprisonnée depuis des années.

que j'ai exposé dans cet hémicycle est simple : j'estime que les crédits publics doivent être modulés en fonction de la charge de service public assumée par les établissements. Élu du département des Hauts-de-Seine, je crois je crois connaître la parlementaire à laquelle vous avez fait référence, monsieur le ministre. Je sais, en effet, que certains établissements privés réalisent un énorme travail pour accueillir des enfants en difficultés. Et figurez-vous que, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, je vote, avec la majorité, les crédits pour les aider.

le ministre, êtes-vous d'accord pour que nous ayons un débat d'orientation avant les calages budgétaires, de façon à prendre un peu plus de temps sur un sujet qui est de la première importance

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Enseignement scolaire », figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits, modifiés.

Cet engagement a été tenu en septembre 2017. Par cet amendement, nous proposons que soit remis un rapport afin d'évaluer l'impact de cette décision.

en tant que rapporteur spécial, mon regard se porte naturellement sur les crédits de la mission. De ce point de vue, elle constitue la vingt-sixième du budget général. Sa dotation progresse de 22 % à périmètre constant et s'élève, à l'issue du vote de l'Assemblée nationale, à 962,3 millions d'euros. Cependant, cette analyse ne saurait suffire, pour trois raisons. La première résulte du caractère central des politiques publiques qu'elle porte. La mission incarne le coeur de notre société : son présent, avec la cohésion sociale portée par les mouvements sportif et associatif ; son avenir, avec le soutien à la jeunesse, et je me réjouis que le Gouvernement poursuive dans la réussite du service civique en 2018, avec un objectif de 150 000 jeunes réalisant une mission l'an prochain. Je m'interroge toutefois sur l'articulation qui sera définie avec le service national voulu par le Président de la République. La deuxième raison s'explique par les perspectives exceptionnelles qui se dessinent à l'horizon. L'attribution récente de la coupe du monde de rugby à la France s'est ajoutée à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ces décisions sont récentes, mais leurs conséquences sont immédiates. Un programme spécifique pour l'Olympiade de 2024 a été créé après le dépôt du projet de loi de finances, doté de 48 millions d'euros de crédits. J'approuve cette démarche, d'ailleurs préconisée par notre collègue Didier Guillaume dans son rapport publié l'année dernière, qui permettra de distinguer les crédits dédiés à cet événement exceptionnel des crédits indispensables au sport pour tous. De même, je note qu'il nous est demandé dans le collectif budgétaire de permettre au comité d'organisation des jeux Olympiques, le COJO, de bénéficier de la garantie de l'État. Cependant, ce comité n'est pas encore constitué et plusieurs interrogations demeurent s'agissant de sa composition et de son fonctionnement. Sa définition doit intervenir avant le 13 février prochain. Sans doute pourrez-vous, madame la ministre, nous donner des précisions à ce sujet. Nous devons donc travailler rapidement sur des dossiers emblématiques, mais aussi coûteux pour nos finances publiques. Dans cette perspective, il est indispensable, madame la ministre, que l'ensemble des documents, en particulier les engagements fiscaux pris par la France auprès du Comité international olympique, nous soit transmis. Je souhaiterais que vous nous assuriez de la pleine collaboration de vos services à ce sujet. Le dispositif national de lutte contre le dopage a favorablement contribué à la réussite française dans ces différents dossiers. Or l'Agence française de lutte contre le dopage doit actuellement faire face à la suspension par l'Agence mondiale antidopage du laboratoire d'analyse de Châtenay-Malabry. Alors que la subvention prévue pour l'AFLD en 2018 est réévaluée afin de prendre en compte l'assèchement de son fonds de roulement, cette suspension pèsera sur les ressources propres de l'agence. Il importe donc de soutenir les capacités françaises de lutte contre le dopage, afin de promouvoir les compétences françaises en la matière et de répondre aux exigences croissantes de l'agence mondiale. La troisième raison pour laquelle une simple analyse fondée sur les crédits ne saurait suffire résulte des modifications opérées par rapport à 2017. Je pense à la suppression de la réserve parlementaire et au Centre national pour le développement du sport,

votre choix s'accompagne d'une atrophie de ses ressources allant au-delà de cette clarification. Le CNDS devra réaliser près de 64 millions d'euros d'économies en 2018. Le compromis proposé par le Gouvernement vise à assurer que le CNDS ne sera plus sollicité pour financer les grands événements sportifs et soutiendra exclusivement le sport dans les territoires. De plus, le Gouvernement s'est engagé à ouvrir près de 30 millions d'euros dans le collectif budgétaire de fin d'année pour le CNDS. Il s'agit d'un choix risqué. Nous estimons absolument primordial de préserver coûte que coûte les moyens alloués au sport dans les territoires. C'est pourquoi le Sénat, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, a relevé le plafond de recettes affectées au CNDS, afin de maintenir le même niveau de ressources en 2018. Ce choix est d'autant plus risqué que, initialement, le Gouvernement entendait ne pas compenser la suppression de la réserve parlementaire. Au-delà des débats sur la réserve elle-même, je tiens à souligner que celle-ci constituait une ressource traditionnelle et essentielle de nombreuses petites associations. En 2017, elle représentait 10 % des crédits destinés à la jeunesse et à la vie associative hors service civique. Une solution de rechange a finalement été définie, consistant à majorer les ressources du fonds de développement de la vie associative de 25 millions d'euros. Cependant, le fonds se concentre pour l'instant sur le soutien à la formation des bénévoles associatifs. De surcroît, ces crédits conduiront à quadrupler la dotation initiale du fonds. Je m'interroge donc naturellement sur les modalités qui seront définies pour l'attribution de ces crédits. Le Gouvernement a précisé qu'un groupe de travail serait constitué pour en décider, afin de permettre un financement dès le début de 2018. En tout état de cause, il importe, madame la ministre, que les petites associations puissent en bénéficier, sans difficultés administratives. La programmation de la mission a donc beaucoup évolué entre le texte initial et le texte transmis par l'Assemblée nationale. Un programme supplémentaire a été créé, et les crédits ont été majorés de plus de 8 %. Compte tenu de ces éléments, et sur ma recommandation, la commission des finances s'est finalement prononcée pour l'adoption des crédits de la mission. je vous remercie Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre commission a donné un avis favorable, avec vigilance, aux crédits du sport dans le projet de loi de finances pour 2018. Notre choix se veut d'abord un signe de confiance dans votre action, madame la ministre, vous qui avez démontré par vos résultats sur les pistes d'escrime votre maîtrise du très haut niveau olympique. Vous savez ce qui est nécessaire pour nos athlètes et votre attachement au développement du sport pour tous illustre votre vision globale des enjeux du sport. Cependant, ce budget n'est pas complètement satisfaisant, car il comporte quelques artifices et surprend par l'absence de moyens véritablement nouveaux pour accompagner nos athlètes. Concernant les artifices, nous avons entendu que la baisse des crédits avait été contenue à 1 % par l'annonce d'un abondement du fonds de roulement du CNDS à hauteur de 27 millions d'euros dans le projet de loi de finances rectificative. Outre que cet engagement doit encore être tenu, il n'apporte pas les mêmes garanties qu'une inscription dans le projet de loi de finances. Le débat budgétaire aurait mérité que l'on puisse mesurer dans la globalité l'effort de la Nation pour le sport. Par ailleurs, la réforme du périmètre d'intervention du CNDS est-elle complète, à la suite de la réduction de moitié de ses moyens et du transfert de ses missions et crédits au programme 219, ou bien faut-il s'attendre à une rebudgétisation supplémentaire ou totale l'année prochaine ? Nous manquons de visibilité sur les intentions à moyen terme du Gouvernement, compte tenu en particulier de l'enjeu que représente la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, même si je sais que ce sera l'un des éléments du débat que vous venez de lancer sur la gouvernance du modèle sportif français. Certes, la préparation de ces jeux semble présenter de nombreuses garanties, dont nous discuterons prochainement à l'occasion du projet de loi olympique. Les critiques émises récemment par la Cour des comptes concernant l'organisation de l'Euro 2016 ne semblent pas de mise pour cet événement,

Ce qui nous inquiète ici, au Sénat, tient moins aux équipements, dont on ne doute pas qu'ils seront livrés à temps, qu'à l'accompagnement de nos athlètes. L'INSEP, l'Institut national du sport, notamment pour construire plusieurs équipements manquants- un dojo de karaté, une salle multisport pour le handball et le volley-ball et un mur d'escalade pour l'épreuve de vitesse. Les crédits d'accompagnement des athlètes de haut niveau doivent nécessairement augmenter pour permettre d'atteindre les objectifs que vous avez fixés, et il existe un risque que cet effort soit tardif et insuffisant. Enfin, l'AFLD est confrontée à des enjeux cruciaux, avec la nécessité de construire rapidement un nouveau laboratoire et de retrouver une activité normale à l'issue de la période de suspension qui devrait s'achever, nous l'espérons, en janvier prochain.

Notre pays aura l'honneur d'organiser les jeux Olympiques en 2024 et la coupe du monde de rugby en 2023. Vous avez raison de considérer que l'héritage doit aussi viser l'augmentation du nombre de pratiquants, mais cela passe par un développement du sport scolaire, du sport en entreprise, du sport santé, etc. Pour répondre véritablement aux enjeux, nous sommes nombreux dans cette assemblée à appeler de nos voeux la mise en chantier rapide d'une loi de programmation budgétaire pour la période 2019-2024, qui seule permettrait au Parlement de jauger et juger l'effort produit par le Gouvernement. La création d'un programme spécifique dédié aux jeux au sein du projet de loi de finances constitue une première étape, mais celui-ci ne tient pas compte aujourd'hui de l'accompagnement des athlètes et des autres aspects que j'ai évoqués- CNDS, AFLD, AFLD, etc. La quasi-stabilité des crédits consacrés au sport a suscité une quasi-unanimité pour faire preuve de bienveillance à l'égard de votre action, madame la ministre. Nous souhaitons que ces encouragements vous permettent, dans les mois qui viennent, de porter « plus vite, plus haut, plus fort » les moyens consacrés au sport dans notre pays.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, les crédits consacrés au programme 163, « Jeunesse et vie associative », se caractérisent par la poursuite de l'effort en matière de service civique et la reconduction des crédits en faveur des autres actions hors réserve parlementaire. Certes, la fin de cette réserve, qui représentait 60 millions d'euros pour les associations en 2017, a une conséquence non négligeable sur leur équilibre financier. Toutefois, vote de l'amendement gouvernemental par l'Assemblée nationale a permis d'abonder le fonds pour le développement de la vie associative de 25 millions d'euros supplémentaires, faisant croître d'autant le budget du programme 163, qui, du coup, n'a jamais été aussi élevé. La commission de la culture ne pouvait donc qu'émettre un avis favorable sur le programme 163, que je réitère aujourd'hui. Cependant, la politique de la jeunesse et de la vie associative ne se limite pas aux crédits de ce programme. Les signaux négatifs envoyés au milieu associatif par le Gouvernement s'accumulent. Déjà touchées par la suppression de la réserve parlementaire, les associations ont été fortement déstabilisées par le changement brutal de politique décidé par le Gouvernement en juillet dernier concernant les contrats aidés. la fixation d'un plafond largement inférieur aux 400 000 contrats aidés enregistrés les années précédentes et du durcissement des critères d'attribution, de nombreuses personnes dont le renouvellement du contrat pour 2017 avait été considéré comme acquis ont dû être licenciées. Les conséquences humaines furent désastreuses, car, il ne faut pas l'oublier, les contrats aidés visent les personnes les plus éloignées de l'emploi et représentent souvent pour elles leur dernier espoir d'insertion sociale ! Du jour au lendemain, elles se sont retrouvées sans perspective. Au-delà de cet aspect humain, le non-renouvellement brutal des contrats aidés remet en cause la pérennité des associations les plus petites et donc les plus fragiles financièrement, qui ont proportionnellement plus recours aux emplois aidés et ne bénéficient pas du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires. En réalité, le Gouvernement ne pourra pas s'exonérer d'une réflexion sur le financement d'activités reconnues utiles socialement, mais qui ne sont pas rentables économiquement, ou alors seulement si elles sont réservées à une minorité. Il est donc temps de reconnaître que la plupart des contrats aidés du secteur non marchand répondent à une demande sociale qu'il conviendrait surtout de financer correctement. Au-delà de la suppression des contrats aidés, d'autres mesures figurant dans le projet de loi de finances pour 2018 risquent de mettre à mal le modèle économique des associations. C'est le cas de la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune

La diminution structurelle des concours financiers de l'État en direction des collectivités territoriales a également un impact négatif sur les associations. Faute de mesures concrètes, le plan de développement pour la vie associative, annoncé par le Premier ministre en début du mois, n'a pas dissipé les inquiétudes. En ce début de quinquennat, il me paraît important d'affirmer que la reconnaissance du secteur associatif, de l'engagement de ses bénévoles et du travail fourni, qui constitue une véritable plus-value sociale, devra se traduire par une valorisation du bénévolat et des financements, notamment au service de de la capacité d'innovation sociale des associations. Ces dernières ont également besoin d'une meilleure visibilité financière et de la poursuite de la simplification des procédures.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en venons maintenant à débattre des crédits accordés à la mission « Sport, jeunesse et vie associative » dans le projet de loi de finances pour 2018. Sur la question sportive, la réduction des crédits de 7 %- soit de 136 millions d'euros -témoigne d'une réelle remise à plat du budget de cette mission, avec une volonté de recentrer les missions du Centre national pour le développement du sport. Nous Nous y sommes sensibles. C'est en effet un effort salutaire dans la perspective de l'équilibre des finances publiques, mais les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, à l'instar d'autres collègues, s'inquiètent du financement des projets d'ores et déjà engagés par le CNDS sur l'année 2018. Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative, le ministre de l'action et des comptes publics a d'ailleurs dû ouvrir une enveloppe supplémentaire de plusieurs dizaines de millions d'euros pour anticiper cette situation. Le CNDS de demain devra davantage s'appuyer sur les missions de proximité, plutôt que de financer la construction de grandes infrastructures sportives. Il faut aller au plus près des Français pour accompagner la pratique sportive. Au sein du programme 219, l'augmentation des crédits de l'action n° 1, Promotion du sport du plus grand nombre, de 35,67 à 89,67 millions d'euros, va dans ce sens et participe de l'effort de mixité sociale. Surtout, ce budget sportif nous invite à anticiper les dépenses à venir dans le cadre de l'accueil de la coupe du monde de rugby, en 2023, et des jeux Olympiques et Paralympiques, en 2024. Ces chiffrages n'ont pas été pris en compte dans le présent budget, puisque la décision d'accueil a été reçue après le bouclage budgétaire. Ce sont deux occasions formidables pour la France, Paris et la région d'Île-de-France. L'adaptation ou la construction des infrastructures sera un sujet épineux de nos débats. En commission, le rapporteur pour avis, notre collègue Jean-Jacques Lozach, a ainsi pointé du doigt une sous-évaluation de certains budgets de rénovation des infrastructures, à l'exemple de la rénovation du Stade de France. thématique « Jeunesse et vie associative », notre groupe salue la pérennisation du dispositif du service civique. Ainsi, 150 000 jeunes pourront participer à une telle mission en 2018, pour un coût de 446,7 millions d'euros. C'est un exercice de citoyenneté et de cohésion nationale qui a fait ses preuves. Son extension sous la forme d'un service universel national, ainsi que l'a proposé le futur Président de la République pendant sa campagne, nous semble donc une bonne mesure, qu'il faudra cependant anticiper sur le plan financier. Nous présenterons, d'ailleurs, un amendement en ce sens au sein de la mission « Défense ». Quant aux initiatives de soutien à la vie associative, nous nous joignons à nos collègues pour saluer l'abondement du Fonds pour le développement de la vie associative de 25 millions d'euros, afin de compenser la suppression « sèche » de la réserve parlementaire. C'est un geste encourageant pour accompagner nos associations, mais il ne faut pas que les efforts de rationalisation conduisent à délaisser ce secteur si important pour le fonctionnement de notre démocratie et de notre société. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement propose un budget équilibré. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera en faveur des crédits de cette mission, tout en appelant à rehausser nos ambitions dans la perspective des grands

la structuration des crédits du sport connaît, au travers de ce projet de loi de finances pour 2018, une évolution importante. Le CNDS et le budget du ministère des sports voient leurs missions et leurs moyens respectifs profondément évoluer. Lors du dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale, l'évolution réelle des crédits dédiés au sport faisait état d'une baisse de 7 %. Toutefois, compte tenu désormais des ajustements annoncés par le Gouvernement dans le collectif budgétaire de fin d'année, ce budget présente une relative stabilité, avec une baisse estimée entre 1 % et 2 % par rapport à l'exercice précédent. En effet, nous avons été nombreux à manifester une profonde inquiétude quant au devenir des projets portés par le CNDS, dont le recentrage des missions sur le sport pour tous doit s'accompagner d'une diminution par deux de ses recettes fiscales affectées. Aussi, le ministère de l'action et des comptes publics a annoncé l'ouverture d'une enveloppe au profit du CNDS de 20 millions d'euros à 30 millions d'euros dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificative. Le groupe du RDSE se félicite de ce rééquilibrage, car le CNDS, fort d'une solide expérience, est un acteur essentiel du soutien au sport dans les territoires. Le sport amateur demeure fortement tributaire de son action. Celui-ci doit déjà pallier la disparition de la réserve parlementaire, qui représentait, en matière de crédits sportifs, 16 millions d'euros par an. Le non-renouvellement de nombreux contrats aidés représente également une difficulté importante à surmonter dans l'animation des clubs amateurs. Enfin, la baisse des dotations allouées aux collectivités a aussi des répercussions très significatives dans le financement du sport pour tous : 72 % du financement public du sport en France sont encore réalisés par nos communes. si le fonds de roulement du CNDS sera porté par la loi de finances rectificative de 49 millions d'euros à, vraisemblablement, 76 millions d'euros l'an prochain, nous resterons attentifs au devenir des projets engagés par le CNDS au-delà de 2018 et dont l'avenir est toujours incertain. Quant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le RDSE juge également indispensable que la mobilisation des moyens requis pour une telle manifestation se fasse au sein d'un programme budgétaire. Le budget du sport, dont le poids financier demeure toujours très modeste dans le budget de la Nation, ne devrait donc pas être amputé dans les années futures du fait de la désignation de Paris et de Marseille, pour le volet nautique, comme villes hôtes. Au sein du programme « Jeunesse et vie associative », nous constatons avec satisfaction que le Gouvernement poursuit l'effort financier précédemment entrepris en faveur du service civique. La reconnaissance des mérites de ce dispositif est désormais largement partagée. Celui-ci devrait permettre à 150 000 jeunes d'effectuer une mission de service civique l'an prochain, contre 130 000 les années précédentes. Un seul regret au-delà des nombreux mérites de ce dispositif, le service civique concentre toujours 83 % des crédits de la politique de la jeunesse et de la vie associative dans notre pays. La vie associative est pourtant fortement affectée par la disparition de la réserve parlementaire. Absolument ! Sur les 146 millions d'euros alloués à la dotation d'action parlementaire, quelque 60 millions d'euros bénéficiaient encore l'an passé aux associations et aux fondations. Le Gouvernement a proposé l'ajout de 25 millions d'euros supplémentaires au Fonds pour le développement de la vie associative. Si nous saluons cet effort budgétaire, nous regrettons toutefois que cette compensation ne soit que partielle, car nous savons tous combien la vitalité du tissu associatif est précieuse pour la cohésion de nos territoires. La non-reconduction d'un grand nombre de contrats aidés vient malheureusement accentuer ces difficultés. L'activité de nombreuses associations s'en est trouvée profondément désorganisée, quand ce n'est pas clairement leur pérennité qui est remise en cause. Nous devons apporter des réponses aux associations qui aspirent à disposer d'un personnel qualifié, mais dont la rentabilité économique ne permet pas de recourir à de tels recrutements sans contrats subventionnés. Personne dans cet hémicycle ne contestera l'utilité sociale et le bénéfice de l'action associative, qui est aujourd'hui privée de plusieurs dizaines de millions d'euros de ressources. Compte tenu du rectificatif budgétaire annoncé en faveur du CNDS, le groupe du RDSE, très attentif aux propositions que pourra prochainement formuler le Gouvernement en faveur du tissu associatif,

Nous ne devons pas décevoir les acteurs sportifs, d'autant plus que la France a obtenu l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, de la coupe du monde de rugby de 2023 et organisera de nombreux autres événements internationaux dans les prochaines années : coupe du monde féminine de football, championnat d'Europe d'athlétisme et d'autres compétitions encore. Dans le même temps, le sport amateur a plus que jamais besoin de soutien pour que son dynamisme demeure et qu'il puisse se développer. que nous soyons à la hauteur de ces objectifs, le Sénat a voté lundi dernier en séance publique, sur notre proposition conjointe avec notre collègue Claude Kern, une hausse de 63,8 millions d'euros du budget du CNDS. Ainsi, nous apportons à la volonté du Gouvernement de soutenir le sport pour tous et le sport amateur les moyens de cette ambition. Très bien ! Au contraire du Gouvernement, le Sénat propose une hausse de 5 % du budget du sport qui, vous le savez, madame la ministre, n'affecterait pas les équilibres budgétaires de l'État. En effet, cet apport n'est simplement dû qu'à la conservation du plafond des taxes sur la Française des jeux affectées au budget du CNDS. Ce mécanisme avait d'ailleurs été proposé par votre majorité à l'Assemblée nationale par le rapporteur général et adopté en commission avant d'être retiré en séance publique. Madame la ministre, vous avez annoncé le lancement de travaux concernant le modèle d'organisation du sport en France. Nous soutenons ces travaux attendus et maintes fois reportés. Mais nous préférons connaître leurs résultats, afin de pouvoir évoquer et débattre du financement du sport dans notre pays. De plus, vous annoncez que le projet de loi de finances rectificative pour 2017 viendra réajuster le budget du CNDS or, nous le savons tous, il s'agit d'un simple remboursement de dettes qui certes sera réalisé en 2018, mais qui n'apportera pas de moyens budgétaires supplémentaires. Ce jeu d'écriture n'est pas à la hauteur de nos débats. Il faut certes renflouer les caisses du CNDS, mais aussi redonner les moyens de son ambition au sport français. C'est là toute la démarche que nous avons entreprise avec nos collègues. Aujourd'hui, le budget que vous nous proposez est ambitieux dans ses objectifs, et nous vous soutiendrons dans les réformes que vous souhaitez mener. Le recentrage des missions du CNDS est, par exemple, attendu depuis de nombreuses années. Toutefois, comme mes collègues l'ont rappelé, le soutien aux investissements locaux doit demeurer un axe important des missions du CNDS. C'est pourquoi les crédits supplémentaires votés par le Sénat permettront aux collectivités locales de continuer à investir et d'être dans leurs projets de rénovation ou de construction des nouveaux équipements, qu'elles ont de plus en plus de mal à financer après les baisses de dotation et la suppression de la réserve parlementaire.

De même, l'introduction par l'Assemblée nationale d'une ligne spécifique pour les jeux Olympiques est un point notable, en termes de transparence et de lisibilité. En effet, il est important que le financement par l'État de cet événement soit totalement transparent, alors que de nombreux scandales ont été mis en avant lors des dernières Olympiades.

De plus, nous savons tous qu'il y a urgence à investir rapidement dans de nouveaux locaux, afin d'offrir les meilleures conditions de travail aux personnels, pour conserver notre expertise dans la lutte contre le dopage et demeurer en tête sur ces questions. Pour conclure, je souhaite évoquer rapidement, car d'autres collègues le feront plus en détail, le budget « Jeunesse et vie associative ». Celui-ci n'est pas satisfaisant : 80 % de son montant est fléché en direction du service civique. Par

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les

Dans ce contexte exceptionnel et mobilisateur, les défis qu'il nous est proposé de relever avec cette mission « Sport, jeunesse et vie associative » passionnent chacun d'entre nous, qui sommes si désireux de voir nos sportifs triompher. Cependant, la réussite sportive de demain se prépare aujourd'hui, en adoptant ce budget, en votant les 348 millions d'euros de crédits du programme 219 « Sport », le développement du « sport pour tous », ainsi que la ligne budgétaire dédiée à la préparation des jeux. Le double objectif des 80 médailles et des 3 millions de licenciés supplémentaires montre l'ambition du Gouvernement dans sa mission essentielle de coordination, d'encadrement et de contrôle de la vie sportive. pour que l'effort consenti soit efficace, il devra être déployé sur l'ensemble du territoire, dans l'hexagone comme dans les outre-mer, dans les grandes aires urbaines comme dans les territoires ruraux et intermédiaires. C'est seulement à ce prix que nous réussirons. En filigrane, la question des infrastructures et des équipements est donc essentielle, parce qu'il en manque ou parce que leur état vétuste les rend impraticables. À cet égard, je tiens à rappeler le constat sans appel dressé en juillet 2016 par l'inspection générale dans un rapport sur les besoins d'équipements sportifs dans les outre-mer. Ceux-ci pâtissent, avec un niveau d'équipement inférieur d'un bon tiers à celui de l'ensemble de la France, d'un net retard aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Madame la ministre, si avez indiqué qu'une enveloppe de 7 millions d'euros à 10 millions d'euros serait dégagée à cet effet, nous aurons besoin d'établir une feuille de route précise sur le développement des équipements sportifs, alors même que le plan de rattrapage activé au 1 janvier 2017 a été interrompu. Vous l'avez dit, la distance ne doit pas nous faire oublier ce que nous devons aux territoires ultramarins et à leurs sportifs- vous-même, vous en êtes le symbole -, mais aussi et surtout ce que nous devons y faire pour reconstruire et encadrer la vitalité de la jeunesse par l'éducation et le sport. Avec ce programme 219, le Gouvernement propose une clarification des interventions en faveur du sport traduisant une volonté de transparence et de simplicité que nous tenons à saluer. Je regrette cependant que nos débats n'aient pas permis de dissiper les craintes du Sénat sur le budget du Centre national pour le développement du sport. Il est vrai que la participation de celui-ci dans la réalisation d'équipements publics de proximité se révèle en pratique très incitative pour les collectivités. Néanmoins, je crois qu'en prévoyant dans la loi de finances rectificative pour 2017 une dotation de 27 millions d'euros permettant au CNDS d'assurer le financement de projets déjà engagés, le Gouvernement a apporté une réponse positive. je rappelle plus globalement que la diminution de 111 millions d'euros est raisonnablement compensée par l'abondement d'autres crédits. La situation est donc moins critique que nous ne le redoutions, même si l'avenir du CNDS reste incertain. En effet, compte tenu des changements de périmètres décidés, les futures missions du centre devront être précisées. J'en viens maintenant au budget consacré à la jeunesse et à la vie associative, qui s'élève à 541 millions d'euros de crédits pour 2018. Ce programme en augmentation poursuit la dynamique du service civique, avec la création de 20 000 postes supplémentaires. Quand on connaît le nombre de volontaires désireux de s'investir et l'expérience positive qu'ils en retirent, ce choix nous paraît intéressant. Dans de nombreux territoires minés par le chômage, il est primordial de travailler le lien social, notamment auprès des jeunes. Le service civique doit leur ouvrir de réelles perspectives professionnelles. Pour cela, il faut veiller à accompagner cette augmentation d'une plus grande variété de missions. Nous le savons, les associations jouent un rôle majeur dans le fonctionnement du service civique, puisqu'elles portent la majorité des postes proposés. Nous ne devons pas être sourds aux vives inquiétudes qu'elles expriment. Elles tiennent parfois à des choses simples. Conscient de leurs difficultés, le Gouvernement a réagi en compensant en partie la suppression de la réserve parlementaire par un abondement à hauteur de 25 millions d'euros supplémentaires sur le Fonds pour le développement de la vie associative. Par ailleurs, il est certain que le changement de politique en matière de contrats aidés affecte les situations déjà fragiles des associations, en particulier les plus petites. Il faudra les accompagner et être vigilants. En ce sens, la mission d'information mise en place par notre commission permettra, j'en suis certain, d'évaluer plus finement l'impact de la réduction des contrats aidés sur le secteur et formuler ainsi des recommandations. Il nous faut donner du souffle aux associations et à leurs bénévoles. Nous savons l'importance du bénévolat dans le sport et plus largement dans le milieu associatif. Nous devons encourager ces femmes et ces hommes qui, par le temps qu'ils consacrent et les initiatives qu'ils prennent, font vivre nos territoires en produisant du lien et de la solidarité. Parce qu'il n'y a pas de réussite sportive sans réussite sociale, l'État doit soutenir sans relâche le monde associatif et sportif. Madame la ministre, les mesures portées par cette mission vont dans le bon sens.

Madame la ministre, l'attribution à la France de l'organisation de la coupe du monde de football féminin en 2019, du monde de rugby masculin en 2023 et des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 met notre pays au défi. Saurons-nous saisir cette chance pour faire de ces événements des moteurs du développement de la pratique sportive pour tous, de porter en avant une forte ambition pour une politique publique d'émancipation par le sport dès l'école et tout au long de la vie ? Si nous n'agissons pas ainsi, nous serons passés à côté de l'essentiel. Atteindre cet objectif suppose pour les cinq années à venir, car c'est maintenant que cela se joue, de changer d'échelle en matière d'ambition sportive dans notre société, donc de changer d'échelle en matière budgétaire. On ne fera pas tout cela avec un budget national du sport qui sera bientôt équivalent au seul budget du PSG ... Le budget que nous examinons rate la première marche. Il est traditionnellement très faible, beaucoup trop faible, mais cette fois il a même été présenté en baisse de 7 %, ce qui est incroyable au lendemain de l'attribution des Même corrigé par le collectif budgétaire et la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale, il demeure en recul, ce qui n'est évidemment pas justifiable à nos yeux. En première ligne de la baisse annoncée des crédits se trouve le Centre national pour le développement du sport, le CNDS. Le recentrage annoncé de ces missions n'explique pas tout. Même en excluant les fonds jusque-là fléchés vers la construction des grandes structures, il manquait près de 50 millions d'euros pour lui permettre d'être à la hauteur de ses missions de promotion du sport pour tous.

La situation est d'autant plus fragile que l'engagement budgétaire des collectivités en faveur du sport, affecté en raison de la baisse des dotations, a eu de lourdes conséquences le monde sportif. Vous affichez, madame la ministre, l'objectif d'une forte augmentation du nombre de licenciés, que nous partageons totalement. Mais,

et aux insuffisances en matière d'équipements sportifs de proximité. Quant au sport scolaire, il reste le grand sinistré de nos politiques publiques en matière de sport. Je soutiens donc la proposition de notre rapporteur Jean-Jacques Lozach que soit mise en chantier une loi de programmation budgétaire. Je propose qu'elle vise un rattrapage massif de ces retards. Je propose également que soit mis en place un observatoire visant à établir un état des lieux de nos installations sportives de proximité, afin que, à partir des inégalités et des retards constatés, on puisse établir un plan de marche national pour la construction de ces équipements et la promotion budgétaire adéquate. Je propose enfin que soit entièrement remise sur le métier une véritable ambition en matière de sport scolaire et universitaire. Alors seulement la perspective des compétitions sportives mondiales que nous allons accueillir pourra-t-elle être le levier qui mobilise le pays pour cet effort national. S'agissant des crédits concernant la jeunesse et la vie associative, ils sont phagocytés par le financement du service civique, qui représente à lui seul plus de 80 % des crédits de la mission. C'est dire que, hors service civique, il n'y a plus de réelle politique publique dans ces domaines Le service civique est un programme intéressant quand il permet à de jeunes volontaires de s'inscrire dans un parcours de citoyenneté. Il peut mettre le pied à l'étrier à des jeunes peu qualifiés, ou pas qualifiés, bien qu'il soit largement utilisé par des jeunes diplômés. dans la réalité, le dispositif sert souvent à permettre aux structures accueillantes de remplacer un emploi qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles ne veulent pas rémunérer. Le service civique devient alors non plus un dispositif d'éducation à la citoyenneté, mais un sas d'entrée dans une vie de précarité pour en quelque sorte une période d'essai sous-rémunérée. Pour le reste, la mise à la diète du monde associatif est criante, notamment en raison de la suppression des emplois aidés, et les politiques en direction de la jeunesse sont réduites à la portion congrue, alors même que les associations ont fait depuis longtemps la preuve de leur utilité en matière de solidarité et de citoyenneté, notamment dans les zones en difficulté Tout cela est pour nous un immense gâchis, surtout un immense manque à gagner, car le sport, la jeunesse, l'éducation populaire- expression qui semble avoir disparu des politiques publiques -appellent de plus grandes ambitions au service de l'émancipation. Le budget rate cette année encore le coche ; nous ne le voterons donc pas. Néanmoins, nous travaillerons, notamment dans la perspective des jeux Olympiques, à une nouvelle ambition de la France pour la jeunesse,

c'est au nom du groupe Union Centriste que je m'adresse à vous afin de faire valoir notre position sur le budget de cette mission, mais aussi de mettre l'accent sur les points de vigilance à propos desquels nous ne manquerons pas d'exercer une attention soutenue. Nous avons suivi l'évolution des crédits de cette mission depuis le dépôt du projet de loi jusqu'aux ajustements qui ont été opérés lors de son passage à l'Assemblée nationale. Nous en prenons acte et, objectivement, nous nous réjouissons de certains signes positifs, non sans garder à l'esprit une perfectibilité non expressément atteinte. Bien évidemment, nous saluons la réorientation des missions du CNDS, qui seront désormais axées sur la proximité. Cette bascule participe d'une volonté de transparence et de simplification, et c'est assurément une bonne chose, parce qu'elle permet au CNDS de renforcer son action en faveur du sport pour tous. Simplement, sous couvert de cette réorientation, son budget a été, de notre point de vue, obéré de façon bien trop importante. De même, la création d'une ligne budgétaire spécifique visant à honorer les engagements souscrits auprès du Comité

Mais pour qu'il soit efficace et pour que le double objectif des 80 médailles et des 3 millions de licenciés supplémentaires soit atteint, il faut que personne, ni rien, ne soit laissé de côté, c'est un défi collectif ! Madame la ministre, pour le remporter, il faut s'en donner les moyens. les moyens. À ce titre, l'abondement du FDVA est un geste fort qu'il convient de saluer. Nous le saluons donc avec les égards qu'il mérite. Cependant, de nombreux points restent en suspens et doivent nous interroger en termes de viabilité, d'efficacité et de pérennisation. Ainsi, le budget du CNDS devait être préservé de manière rationnelle et pragmatique. C'est bien ce que nous avons voulu porter, notamment avec mon collègue Michel Savin, par le truchement de cet amendement soutenu par de très nombreux cosignataires, que je tiens tout particulièrement à remercier ici, adopté lundi dernier et qui rétablit 63,8 millions d'euros au regard des 137 millions d'euros de ressources amputées sur les taxes affectées au CNDS. Le CNDS, nous le savons tous, possède une expertise unique sur la question du sport pour tous, qui est en l'occurrence une volonté revendiquée par le Gouvernement dans sa feuille de route. Dès lors, avec la baisse significative de ses ressources et les économies qui lui sont imposées, ce sont le sport amateur et le sport pour tous qui pourraient en pâtir. Encore une fois, il est important de saluer le geste du Gouvernement pour 2017 ; cependant, l'importance du CNDS est telle qu'il nous a semblé primordial de pérenniser son budget pour 2018. Ce budget, qui ne cesse de se réduire depuis des années, affecte fortement, par effet de ricochet, les subventions accordées par les collectivités locales, qui sont tout de même la première source de financement du sport en France. Le rôle des collectivités locales en matière de développement des pratiques sportives et de soutien à leur exercice devrait pourtant se voir pleinement reconnu. Les atteintes diverses et variées portées au budget des collectivités ont déjà provoqué au cours des dernières années une baisse inévitable des soutiens aux associations et des investissements dans la construction et l'entretien des équipements sportifs. Ces ressources ont encore été amoindries au travers de plusieurs décisions arbitrées par le Gouvernement, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, telles que la fin des contrats aidés et la suppression de la réserve parlementaire. la majeure partie du financement public du sport en France s'opère les communes, c'est un fait. Se présente ainsi une menace réelle pour le tissu associatif sportif. Nous sommes en attente de réponses concrètes du Gouvernement sur cette question centrale. Quelle que soit la beauté du geste, l'abondement du FDVA ne saurait compenser le déficit de ressources dont souffrent les associations sportives à cause de la suppression de la réserve parlementaire. La baisse du nombre de contrats aidés ne risque-t-elle pas de fragiliser encore un peu plus le secteur associatif, donc la vie associative, ciment- faut-il le rappeler ? -de nos territoires et de la cohésion sociale ? de la cohésion sociale ? C'est dans un esprit de clarification que nous avons décidé de confier, au sein de la commission de la culture, une mission d'information sur l'impact de la réduction des contrats aidés à nos collègues Alain Dufaut et Jacques-Bernard Magner. De ce tissu associatif, il faudra travailler la trame de façon cohérente, en impliquant toutes les parties prenantes autour des priorités définies à l'échelon tant national que local, en fonction des besoins spécifiques des territoires. Par ailleurs, nous devons questionner le Gouvernement quant à sa position concernant le bénévolat, car, nous le savons, le FDVA y oeuvre de façon importante, notamment dans la formation des bénévoles, si précieux pour nos associations. Enfin, je me dois d'évoquer le suivi des athlètes. Quelques évolutions sont appréciables, mais la question de leur accompagnement reste entière. On sait que les résultats aux sont fortement dépendants de l'investissement public. Dès lors, il faut espérer que cet investissement commencera d'être réalisé dès 2019, n'est-ce pas ? J'en arrive au terme de mon intervention. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous approuvons et voterons les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », mais tous ces points de vigilance que je viens de pointer nous tiennent en haleine. Sur chacun d'eux, nous ne manquerons pas d'exercer notre droit de regard, sans nous dispenser

très important pour nous. Bien évidemment, nous voterons cette mission. Je ne reviens pas sur la fin des contrats aidés, que nous trouvons beaucoup trop brutale. Si l'on peut comprendre la philosophie qui vous anime, même si on ne la partage pas, on ne peut admettre que, du jour au lendemain, des jeunes se retrouvent sans rien. Surtout, au moment où il faut structurer une vie sociale, un vivre ensemble, les associations ne disposent plus de ces moyens qui leur étaient essentiels. Or elles n'ont pas elles-mêmes les moyens de remplacer ces contrats aidés par des emplois pérennes. En outre,

Il ne peut pas être une coquille vide ; il faudra avancer des propositions, parce que le sport de haut niveau et de très haut niveau ne se nourrit que du sport pour tous. Tout à l'heure, Pierre Laurent parlait du sport scolaire ; ce sont là des valeurs qui doivent aller

Madame la présidente, madame la présidente de la commission, cher Jean-Michel Blanquer, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le budget que je viens vous présenter est un budget de transformation audacieuse. Ce budget nous invite à remettre en cause nos habitudes, nos routines, à repenser profondément notre modèle d'intervention publique. Il permettra, monsieur Pierre Laurent, de changer d'échelle pour le sport. En effet, la dépense publique allouée au sport en France est l'une des plus élevées de l'Union européenne. Or nos résultats ne sont pas toujours à la hauteur, Or nos résultats ne sont pas toujours à la hauteur, et même ils n'y sont pas du tout. Désormais, le ministère des sports doit pleinement s'adapter aux nouvelles pratiques de nos concitoyens, sans jamais perdre de vue ses missions essentielles

enfin réinterroger la haute performance, sur le fondement des propositions qui seront formulées par Claude Onesta. Concrètement, nous augmentons les moyens alloués aux fédérations sportives, grâce à une enveloppe de 3 millions d'euros supplémentaires, afin de porter ces moyens à 76 millions d'euros. Parallèlement, nous prévoyons un investissement exceptionnel de 1,5 million d'euros pour le sport paralympique, afin de préparer au mieux les futures échéances. Nous augmentons de 600 000 euros le soutien personnalisé aux sportifs de haut niveau, soit une enveloppe de plus de 10 millions d'euros. Enfin, recevoir les jeux Olympiques et Paralympiques est une formidable chance économique et sociale. sociale. Vous le savez, nous avons acté la création d'un programme budgétaire pour les Jeux de 2024. C'est une garantie, monsieur Kern, d'un budget maîtrisé.

Je conduis une politique déterminée pour le sport bien-être, le sport santé, le sport sur tous les territoires et pour tous les publics, bref, vous l'avez compris, pour le sport partout, pour tous et tout au long de la vie. Mon but est d'attirer trois millions de pratiquants en plus. Ce budget est la première étape pour remplir cet objectif ; c'est pourquoi nous procédons à un changement de périmètre entre le Centre L'objectif est de rendre l'action du CNDS plus efficace ; celui-ci devient l'opérateur du sport pour tous et le promoteur de l'innovation sociale, fort du plan Héritage 2024, qui sera doté d'une enveloppe de 20 millions d'euros. Ce dispositif sera revisité en 2018, au bénéfice des projets de transformation sociale. Le CNDS continuera de financer les équipements sportifs de proximité à l'échelon territorial, mais ses ressources seront dédiées aux équipements sportifs innovants.

Ce budget est dédié à toutes les pratiques sportives. Or, pour avoir trois millions de pratiquants en plus, il sera impératif de mieux connaître les attentes des Français et d'identifier les ressorts qui inciteront ceux qui ne pratiquent pas encore. Pour ce faire, nous consacrerons 1 million d'euros à des missions d'expertise majoritairement orientées vers le sport pour tous. En outre, mon ministère prend toute sa place dans les discussions interministérielles.

Le sport pour tous, mais aussi partout. Vous l'avez rappelé, monsieur Karam, nous devons beaucoup aux outre-mer ; c'est pourquoi nous dégagerons une enveloppe de 7 millions d'euros à 10 millions d'euros pour les équipements sportifs d'outre-mer et de Corse. Par ailleurs, nous recherchons un effet levier grâce à l'appui technique de l'AFD, Enfin, l'intégrité dans le sport est une priorité du Gouvernement. Le budget de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD, bénéficie d'une augmentation de 10 % de son budget annuel. Nous engageons d'ailleurs une étude de programmation pour un laboratoire adapté aux jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, mes priorités pour le budget 2018. ce qui le concerne, le programme « Jeunesse et vie associative », porté par mon collègue Jean-Michel Blanquer, que je salue, s'articule autour de trois priorités. La première est l'accompagnement vers l'autonomie ; c'est l'objet de notre action pour la jeunesse et l'éducation populaire. L'information, la mobilité internationale et l'accès de tous les jeunes à des loisirs de qualité sont confortés par le présent budget, qui y consacre 25 millions d'euros. Les associations du secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire seront financées à hauteur de 52 millions d'euros, dont 31 millions d'euros le FONJEP, qui soutient plus de 5 000 emplois, et 21 millions d'euros destinés aux associations agréées à l'échelon national ou local. Deuxième priorité, le développement de l'engagement dans la vie associative. À périmètre constant, l'appui au développement de la vie associative progressera de 10 millions

Je souligne que, au-delà de ce soutien transversal aux associations, l'État dans son ensemble contribue fortement au développement de la vie associative, différents dispositifs fiscaux, dont le total rattaché au présent programme 163 dépasse 2,7 milliards d'euros Cet effort sera encore renforcé en 2019 par une réduction pérenne des cotisations patronales bénéficiant au monde associatif à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen en séance publique des crédits de cette mission à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé un amendement visant à relever de 25 millions d'euros les crédits du programme 163, « Jeunesse et vie associative ». Cet amendement a été adopté à l'unanimité. Il s'agit ainsi de compenser, selon des modalités d'attribution renouvelées, la diminution de crédits ouverts au bénéfice du tissu associatif après la suppression de la réserve parlementaire. Ces crédits supplémentaires abonderont le Fonds de développement de la vie associative et, comme il est précisé dans l'amendement du Gouvernement, ces 25 millions d'euros de crédits supplémentaires s'adresseront en priorité

le service civique. Celui-ci s'inscrit dans la continuité de la politique éducative, un quart des volontaires étant peu ou non diplômés. Ce succès se traduit dans les chiffres, en hausse constante depuis maintenant sept ans. Après 92 000 personnes en 2016, ce sont environ 130 000 volontaires qui auront bénéficié du dispositif en 2017. Le budget pour 2018 consacre les moyens accordés au service civique. La cible est fixée à 150 000 volontaires. Les crédits sont augmentés de 63 millions d'euros, pour atteindre 448 millions d'euros. Cette action déterminée sera complétée et encore renforcée par l'engagement du Président de la République de mettre en place un service national universel, dont les modalités sont en cours d'élaboration. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre soutien ; je ne doute pas que nous partageons les mêmes objectifs. Nous